monsieur le président.

le rapporteur général questionnait le Gouvernement : il lui demandait de bien vouloir nous expliquer en quoi les bitcoins, l'or, les diamants et les actions chinoises participaient de l'investissement productif.

Gérald Darmanin a eu l'occasion de répondre ce matin à la question que vous posez. Vous connaissez, comme moi, le caractère novateur des bitcoins. Nous aurons l'occasion d'en reparler à de multiples reprises. Dans l'attente, nous sommes extrêmement favorables au maintien des équilibres sur l'IFI. C'est la raison pour laquelle je serai défavorable à tous les amendements qui visent à dénaturer cet

nous ne pouvons pas nous désintéresser, l'augmentation du plafond de la réduction d'impôt, plutôt que de son taux, permet de maximiser l'effet déclencheur et de minimiser le coût budgétaire de la mesure, tout en limitant ses effets d'aubaine.

Depuis la suppression de l'ISF, nous constatons une chute de 40 % de la collecte de capital pour ces entreprises, qui réalisent un travail très important. En effet, elles parviennent à produire

l'amendement n° I-705. Cet amendement vise à modifier les modalités de calcul du mécanisme de plafonnement de l'IFI en fonction des revenus pour permettre aux contribuables plafonnés de bénéficier de la réduction d'impôt au titre des dons.

pour le calcul de l'imposition de sa plus-value. La suppression de ces abattements pénalise largement les détenteurs de titres émis par de jeunes PME. En effet, les intéressés pouvaient bénéficier d'un abattement susceptible de s'élever jusqu'à 85 % pour une durée supérieure à huit ans, dans le cadre du régime d'abattement renforcé. Cette suppression n'est pas cohérente avec l'esprit de la réforme de la fiscalité du capital engagée en 2018, dans la mesure où elle décourage la création d'entreprise. Les abattements pour durée de détention doivent donc s'appliquer aux plus-values de cession des titres éligibles, quelle que soit la date de souscription ou d'achat.

nous, ces amendements tendent à généraliser un système complexe, applicable dans le cadre d'une clause de sauvegarde clairement encadrée, et à contre-courant des objectifs de lisibilité et de simplification.

présenter l'amendement n° I-706. Si l'instauration du PFU se justifiait par l'amélioration de la lisibilité du système d'imposition des revenus mobiliers, elle a fait l'objet de critiques quant aux possibilités d'optimisation fiscale désormais ouvertes

La baisse annoncée du taux d'impôt sur les sociétés devrait augmenter le différentiel de taxation entre les revenus du capital et les revenus du travail résultant de l'instauration du PFU. Dans cette perspective, notre amendement vise à instaurer une clause anti-abus, que la Haute Assemblée a déjà adoptée lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018. Pour les salariés, dirigeants et cadres possédant plus de 10 % des droits de vote d'une société, le bénéfice du PFU serait plafonné à la fraction du rendement en capital considéré comme normal, c'est-à-dire dans la limite de 10 % du capital investi. Cette option, retenue notamment par la Suède, s'inspire d'une disposition existant déjà pour le traitement des titres logés dans un plan d'épargne en actions ou pour les cotisations des gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée. Les produits et plus-values ne bénéficient de l'exonération d'impôt que dans la limite de 10 % du montant des placements. Dans le cas des travailleurs indépendants, le bénéfice du PFU serait plafonné à la part du revenu n'excédant pas 10 % du capital social et du compte courant d'associé.

Toutefois- nous le savons -, nous sommes dans un contexte économique particulier, avec des taux bas et une épargne majoritairement investie dans des contrats en euros à capital garanti. Cette situation n'est ni pérenne pour le secteur de l'assurance, ni efficace pour l'économie, ni bénéfique pour les Français. Les études menées auprès des gestionnaires d'actifs montrent que la réforme de l'IFI a pour effet de diminuer l'investissement dans l'immobilier et de renforcer l'investissement dans des supports de type « unités de compte Parmi les mesures de la loi Pacte relatives à l'assurance vie, l'article visé par notre amendement cherche à rendre plus attractifs les contrats euro-croissance, ou fonds diversifiés.

Les établissements des secteurs social et médico-social remplissent, vous en conviendrez, des missions d'intérêt général. Toutefois, ils sont assujettis à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances.

Avec cet amendement, nous proposons de généraliser le recours au taux moyen d'imposition avec déclaration mondiale, afin que le recours à la règle des 20 % d'imposition devienne l'exception. Nous souhaitons que ce taux moyen d'imposition, retenu

métropolitaine ! Il serait possible, et utile, de se fonder sur un système d'imposition plus simple et plus équitable : il ne s'agit pas de nier les particularités de nos concitoyens résidant à l'étranger, mais d'améliorer le dispositif existant.

qu'en cas de contrôle. Cette solution permettrait de simplifier l'accès au taux moyen, afin que nos concitoyens ayant des revenus faibles ou modestes ne soient pas sommés d'acquitter l'impôt dès le premier euro.

Le Gouvernement ne peut tout simplement pas, sous prétexte de conséquences néfastes et prévisibles sur les contribuables français, reporter d'un an- année importante, certes, parce qu'électorale -l'échéance de sa mise en place.

Il faut bloquer le projet de réforme, tel qu'il est proposé, en adoptant cet amendement. Nous sommes totalement opposés à cette réforme fiscale et souhaitons purement et simplement que ses règles ne soient jamais appliquées, tant elles sont discriminantes envers nos concitoyens établis hors de France. le coeur de cette réforme ? Si elle entrait en vigueur, une personne qui gagne 27 000 euros par an, soit un peu plus 2 000 euros par mois, serait imposée à 20 % dès le premier euro. Il s'agit là de revenus modestes, dans un grand nombre de pays où le coût de la vie est très élevé. De plus, les Français établis hors de France ne bénéficieraient pas du système fiscal progressif- par tranches sur les premiers seuils d'imposition applicable aux Français de métropole. Nous prônons donc le rétablissement d'une imposition progressive plus proche du droit commun. Mais nous tenons tout de même compte des particularités des Français de l'étranger. La progressivité de l'impôt relève de la justice sociale. Rappelons que les Français de l'étranger n'ont pas peur de déclarer leurs revenus mondiaux et qu'ils s'acquittent de leurs obligations fiscales. Au lieu de faire converger les systèmes fiscaux, la réforme proposée introduit une différence de traitement et complexifie un

pour étudier l'ensemble des effets de cette réforme de la fiscalité des non-résidents.

Les cris d'orfraie que nous avons entendus de la part des Français de l'étranger sont donc parfaitement justifiés, dans la mesure où ils ont découvert que, d'une année sur l'autre, on avait augmenté leurs impôts de 50 %.

du Gouvernement ? Pour les contribuables non résidents ayant les revenus les plus faibles, il nous semble que le souci d'équité fiscale qui anime les intervenants est déjà pleinement satisfait par le dispositif actuel, lequel permet, sur demande, de tenir compte du taux d'imposition moyen du contribuable non résident, calculé sur la base de ses revenus mondiaux. Votre souci de simplification de la production des pièces justificatives est également satisfait. Généraliser le taux moyen alourdirait les obligations déclaratives des contribuables non résidents en les obligeant à déclarer l'ensemble de leurs revenus mondiaux, quand bien même ils n'y auraient pas intérêt ou ne le souhaiteraient pas. Par ailleurs, vous le savez, l'article 2 propose un moratoire d'un an pour les mesures concernant la retenue à la source des non-résidents, ainsi que la remise d'un rapport au Parlement avant le 1 juin afin que les décisions nécessaires puissent

Dans un récent reportage diffusé sur France 2, le ministre Gérald Darmanin affirmait faire en sorte de « rendre plus riches les plus pauvres », et critiquait le président de la commission des finances, notre collègue Vincent Éblé, en affirmant que les socialistes voulaient « rendre plus pauvres les plus riches

les riches plus riches. L'enquête de l'Insee publiée cette semaine prouve d'ailleurs que les mesures socio-fiscales que vous avez mises en place ont favorisé les 10 % de Français les plus aisés, le plus bel exemple de votre générosité étant l'abandon de l'ISF, mis en place par Michel Rocard, entraînant tout de même une perte de recettes fiscales d'environ 3,2 milliards par an. Nous avons très largement débattu de ce point ce matin. Concernant la réforme fiscale pour les Français de l'étranger, il me semble utile de rappeler que les députés de la majorité présidentielle l'ont tous votée il y a un an, mais que, conscients de leur erreur, ils en ont demandé la suppression devant la représentation nationale. Malheureusement, ils n'ont obtenu que le report d'un an de sa mise en oeuvre, alors que

Or les élections consulaires, qui vont désigner les élus de proximité qui représenteront nos trois millions de compatriotes, se tiendront les 16 et 17 mai 2020. L'objet du présent amendement est donc d'avancer la date de remise de ce rapport au 1 mai 2020, dans un souci de transparence vis-à-vis des électeurs établis hors de France, afin de leur garantir une information pleine et entière sur le contenu de cette réforme. Comme mes collègues sénateurs socialistes représentant les Français établis hors de France, je suis attachée à une fiscalité juste et égale entre Français vivant à l'étranger et Français de métropole, c'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous demandons de voter cet amendement.

vise à demander la mise en place d'un simulateur, comme il en existe pour toutes les feuilles d'impôts en France, qui vous permet de connaître directement le niveau d'impôts que vous aurez à payer. Nous, nous n'en avons pas

calcul, car celui-ci repose sur l'application du taux minimum ou sur l'application du taux moyen en cas de déclaration des revenus mondiaux. L'administration va enrichir la documentation disponible pour permettre aux usagers d'utiliser le simulateur actuel pour déterminer si l'option du recours au taux moyen et de la déclaration des revenus mondiaux leur est favorable. D'ores et déjà, mais cela devra être précisé sur le simulateur, lorsque l'usager demande l'application du taux moyen d'imposition, celui-ci est appliqué uniquement s'il est plus favorable que l'application du taux minimum. Ainsi, un usager ayant opté pour l'application du taux moyen et pour lequel le taux minimum s'avère plus favorable se voit automatiquement appliquer ce dernier taux. La demande d'option pour le taux moyen est donc avantageuse pour l'usager dans tous les cas, dès lors qu'il procède ainsi sur le simulateur. Il faut que nous puissions mettre en place des actions de communication pour permettre aux non-résidents de savoir que le fait de demander l'application du taux moyen sur le simulateur est la meilleure façon d'être renseigné, puisque,, l'option la

car les réformes inscrites dans l'article 13 de la loi de finances pour 2019 ont été adoptées sans étude d'impact préalable. Nombre de nos compatriotes nous en décrivent

Cet embrouillamini a suscité des inquiétudes et des protestations bien légitimes chez nombre de nos compatriotes qui nous en ont saisis. Dans l'incitation à déclarer les revenus mondiaux, certains ont vu une orientation vers un impôt sur la nationalité. Les protestations sont telles que la majorité de l'Assemblée nationale a dû proposer un moratoire partiel. Le législateur est ainsi contraint de revenir sur des mesures votées il y a un an, dont le Gouvernement avait célébré les vertus. Le Parlement ne serait pas dans l'obligation de revenir sur ces réformes improvisées s'il avait été mis en mesure d'en apprécier les effets par une véritable étude d'impact communiquée en temps opportun Le rapport prévu par l'Assemblée nationale en matière de fiscalité des Français de l'étranger tend donc à faire ce qui n'a pas été fait en novembre-décembre 2018 : une étude exhaustive des réformes engagées. Notre amendement vise à ce que l'information du Parlement porte sur toutes les conséquences de l'article 13 de la loi de finances pour 2019, car le Parlement a droit à une information complète, une comparaison effective et chiffrée des effets de la législation antérieure et du régime adopté en 2019, y compris les effets résultant du moratoire partiel voté par la majorité de l'Assemblée nationale et de l'application du prélèvement à la source sans les déductions, réductions de charge et exonérations dont bénéficient nos compatriotes résidents. Nous proposons donc d'ajouter

? Je demande le retrait de cet amendement, car le rapport sur la fiscalité des non-résidents, qui sera remis avant le 1 juin 2020, étudiera l'impact des mesures législatives adoptées récemment, notamment de la suppression de la retenue à la source spécifique partiellement libératoire de l'article 182 A du CGI, ainsi que la question de l'application aux non-résidents de la décote. Vous avez évoqué d'autres sujets dans votre intervention, monsieur le sénateur, qui seront intégrés à ce rapport, engagement est pris au banc en ce sens. Je mets aux

Le Gleut. Il s'agit d'un amendement de précision. Les auteurs de la réforme de 2019 ont parlé d'assimilation du régime fiscal sur les revenus de source française entre résidents et non-résidents, mais une telle assimilation serait discriminatoire sans l'application des mêmes règles en matière de déductions, de crédits d'impôt, d'exonérations et de quotient familial que celles qui sont accordées aux contribuables résidents. La question se pose en particulier en matière d'avantages accordés pour l'acquisition d'un logement ou pour une rénovation énergétique. Le Parlement doit être, par conséquent, complètement informé sur les conséquences de la réforme de 2019 dans ce domaine, avant la cessation du moratoire.

M. Ronan Le Gleut. Notre amendement vise à ce que l'information du Parlement porte sur toutes les conséquences de l'article 13 de la loi de finances pour 2019. Le Parlement a droit à une information complète, en particulier à une comparaison effective et chiffrée des effets de la législation antérieure et du régime adopté en 2019, y compris les effets résultant du moratoire partiel voté par la majorité de l'Assemblée nationale. Il s'agit également d'obtenir des informations sur le passage du moratoire décidé par le présent article au nouveau régime applicable en vertu de l'article 2 voté par l'Assemblée nationale après la cessation dudit moratoire.

Pour les non-résidents, il existe deux difficultés majeures. Tout d'abord, en cas de trop-perçu, ou même de simple présomption de trop-perçu de la part du contribuable non résident, c'est à ce dernier de faire une demande auprès de l'administration fiscale pour signaler qu'il a peut-être payé trop d'impôt sur le revenu. D'autre part, en cas de trop-perçu, le remboursement se fait par chèque, et non par voie dématérialisée, ce qui occasionne de nombreuses pertes de courriers et oblige les contribuables à faire des démarches complexes et longues pour faire valoir leur bon droit. Ces situations sont anormales et constituent une rupture d'égalité entre citoyens : pour les résidents, la procédure est différente, puisque le remboursement par virement

! Je persiste à penser qu'il est juste. Il concerne la déductibilité de certaines charges, comme cela existe en France,

l'avis de la commission ?

suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire aux contribuables établis dans les États membres de l'Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leurs revenus mondiaux imposables. Il s'agit souvent de pensionnés.

monsieur le ministre

Le présent amendement a pour objet d'accorder aux contribuables une réduction d'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants

ayant été pénalisé par la disparition de l'ISF, mais surtout du dispositif ISF-PME, les lois de finances pour 2018 et 2019 ont revalorisé le dispositif IR-PME, en portant la déduction fiscale de 18 % à 25 % du montant investi dans les entreprises solidaires. Malheureusement, ce nouveau dispositif n'est pas entré en vigueur, à cause d'un risque de non-conformité aux règles européennes. Ce très long amendement vise à trouver une solution

le montant annuel des dépenses ne pouvant excéder 10 000 euros par personne hébergée. Or les sommes engagées au titre de la dépendance peuvent s'avérer particulièrement élevées. C'est pourquoi M. Chaize propose de relever le plafond de 10 000 à 20 000 euros, en sorte que la réduction d'impôt soit moins déconnectée des montants effectivement engagés.

l'augmentation importante de cet impôt en 2011, dans de nombreux cas, les personnes qui ne pouvaient pas s'acquitter des droits se sont maintenues en indivision, donc dans une situation juridique peu confortable pour elles. Il en va de même en cas de succession ou lors de la vente d'un immeuble acheté en indivision par deux partenaires de PACS ou deux concubins.

de la fiscalité. Mais comme je l'ai dit, nous considérons que le régime actuel est équilibré : en particulier, de nombreuses dispositions favorisent les transmissions en ligne, et 82 % des transmissions sont exonérées de droits de succession. J'ai eu l'occasion, lors de l'examen de la proposition de loi sur les donations et les successions qui avait été déposée par le groupe socialiste,

millions de salariés travaillant dans ces entreprises industrielles seront concernés par ce fait économique majeur. Malgré l'instauration du pacte Dutreil en 2003, la transmission en France reste plus coûteuse que chez nos principaux partenaires européens- son coût est de 11 % en France, contre moins de 5 % en moyenne en Europe. Acquitté par l'entreprise au prix d'une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoût de la transmission en France prive les PME et les ETI de ressources pour grandir, investir, innover et recruter. Pour y remédier, et face à l'urgence économique que constitue la transmission dans les prochaines années, la délégation sénatoriale aux entreprises a sonné l'alarme dans un rapport d'information de février 2017 qui a donné lieu à l'adoption, par le Sénat, le 7 juin 2018, de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise déposée par MM. Claude Nougein et Michel Vaspart, Mme Élisabeth Lamure, M. Bruno Retailleau et de nombreux collègues. Un bon nombre des dispositions de cette loi ont été intégrées dans le projet de loi de finances pour 2019 puis définitivement adoptées, contribuant ainsi à la modernisation du dispositif. Toutefois, l'article 8 prévoyait une extension des conditions de donation, non reprise lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019 : l'exonération partielle par suite d'une donation, actuellement réservée au seul cas où les donataires sont des descendants du donateur, aurait été étendue à tous les ayants cause, sous la seule condition que le donataire puisse poursuivre l'engagement individuel. Une telle possibilité est déjà ouverte pendant la phase d'engagement collectif. Le présent amendement a pour objet de reprendre cette extension, adoptée par le Sénat le 7 juin 2018, car il apparaît essentiel que la transmission d'entreprises

Cette mesure permettra d'ouvrir davantage le dispositif, et donc, d'augmenter les chances de reprise des entreprises dans les années à venir.

visant à le renforcer. Nous considérons que l'équilibre que nous avons trouvé il y a maintenant un peu plus de douze mois doit être préservé. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons aux amendements visant à le modifier. Par ailleurs, nous considérons que la disposition

: La parole est à M. Franck Menonville. Cet amendement vise à favoriser l'ancrage territorial des entreprises implantées en France et, tout particulièrement, celles dont la croissance s'inscrit dans le long terme.

En cas de non-respect de cette durée de détention, les droits de mutation seraient acquittés de la durée de conservation.

Toujours pour favoriser la transmission des petites et moyennes entreprises, ma collègue Élisabeth Lamure propose de compléter l'amendement précédemment adopté par le Sénat et d'instaurer un pacte de très long terme, qui vise à aligner la France sur la moyenne européenne en matière de transmission. L'amendement tend à introduire un nouvel article

Cette mesure servirait un triple objectif d'intérêt général : tout d'abord, la stabilité de long terme des actionnariats, laquelle contribue à la pérennité du développement des entreprises et au maintien des centres de décision et de production sur le sol français

Ainsi, la valeur des biens et droits hérités en ligne directe depuis moins de dix ans viendrait en déduction de l'actif successoral. La valeur déclarée serait réduite du montant des droits de succession acquittés à la suite du premier décès, ce qui conduirait nécessairement à prendre en compte

est défavorable aux deux amendements, car le système actuel comporte déjà des dispositions très favorables aux transmissions en ligne directe. De fait, seuls les contribuables les plus aisés profiteraient de telles mesures, lesquelles contreviendraient au principe de l'imposition en fonction du degré de parenté, en aboutissant par exemple à ce qu'un héritier tiers

Ce montant est identique à celui qui vaut pour les successions proprement dites. Un abattement de 100 000 euros, en lieu et place de celui de 152 000 euros, n'aura d'incidence que sur un très faible nombre de contrats d'assurance vie, comme le montrent bien les chiffres publiés en 2017, les choses n'ayant que marginalement évolué depuis

transactions financières a été créée après la survenue de la crise de 2008 pour que le secteur bancaire, ayant largement bénéficié de l'explosion des flux financiers internationaux, mais ayant été sauvé par la puissance publique pendant la crise, participe à la lutte contre l'extrême pauvreté et les changements climatiques.

Dans un contexte de désengagement des États-Unis en matière de lutte contre le changement climatique, la hausse de ces ressources concourrait à la traduction en faits des ambitions affichées par le Gouvernement.

Ces fonds ont pour objet de contribuer à la pérennité économique des sociétés transmises. Ils pourront par ailleurs financer des oeuvres ou missions d'intérêt général. Le présent amendement a pour objet de préciser le traitement fiscal des opérations de constitution de ces fonds. ces fonds. Une éventuelle plus-value réalisée par l'entreprise donatrice serait mise en sursis jusqu'à la cession des titres transmis par le fonds de pérennité bénéficiaire de la transmission. Dans cette situation, la plus-value, ou moins-value, est prise en compte dans le résultat fiscal du fonds de pérennité lorsque celui-ci cède ultérieurement les titres, par exemple lors de sa dissolution. Le calcul de cette plus-value, ou moins-value, s'effectuera alors à partir de la valeur d'origine des titres dans les écritures fiscales de l'entreprise ayant procédé à la transmission.

Actuellement, les propriétaires qui vendent leurs biens à un établissement public foncier local (EPFL) disposent d'une exonération des plus-values immobilières, sous réserve que l'établissement public foncier rétrocède le bien dans un délai de trois ans à un organisme de logement social. À défaut de respecter cette condition de délai, l'EPFL se trouve redevable du paiement de la plus-value. Dans la pratique, cette disposition se révèle souvent inapplicable,

Le I du présent amendement a pour objet d'atténuer l'effet de seuil résultant de l'application de ce dispositif en permettant aux impatriés ayant résidé seulement trois ans à l'étranger de bénéficier du régime d'exonération forfaitaire de 30 %, non pas sur huit ans, mais sur quatre L'objectif est d'offrir un palier en proposant un avantage réduit dans le temps, de sorte à limiter l'incidence du facteur fiscal sur les décisions de mobilité et de renforcer la capacité de recrutement des entreprises françaises. Le II gage cette mesure sur la taxe sur les sodas. Quel

Le présent amendement vise à rétablir le système d'imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, système plus communément appelé et antérieur à 2019. Ce dispositif de lutte contre l'évasion fiscale, issu de la présidence de Nicolas Sarkozy- monsieur le ministre, vous devez y être sensible,

Des filières renommées et fortement exportatrices font face à des pertes importantes et à la spéculation d'investisseurs étrangers. La spéculation sur le foncier agricole fait en effet partie des causes structurelles de la crise. De plus en plus de terrains détenus ou exploités dans le cadre familial, porteur de valeurs et de savoir-faire uniques, sont ainsi menacés de reprise par des investisseurs, souvent étrangers, suivant une logique purement financière. À terme, cela représente un risque de perte de savoir-faire, de puissance économique, mais aussi de souveraineté. Cet amendement tend à répondre à ces difficultés en exonérant de droits de mutation, d'une part, les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole, d'autre part, celles intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole. Afin d'apporter des garanties nécessaires de la part des propriétaires ou exploitants dans la stabilité et la pérennité de leur engagement, conditions strictes devront être respectées, en particulier une durée de conservation de dix-huit ans minimum dans le patrimoine du repreneur, sous peine de se voir appliquer des rappels et sanctions. Par ailleurs, il est proposé une exonération de l'impôt sur la fortune immobilière

fin ! Cet amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions, lorsque les héritiers s'engagent à ne pas vendre les biens reçus et à les laisser affectés à l'exploitation familiale pendant une durée d'au moins ans. La fiscalité applicable à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes incite les propriétaires à repousser les transmissions en raison de la valeur élevée de ces biens. Ainsi, lorsque s'ouvre une succession, les héritiers sont incités ou contraints à vendre les biens, compte tenu des droits à payer, avec des risques pour la survie même de l'exploitation familiale. Les biens loués par bail à long terme bénéficient d'une exonération partielle à condition de conserver les biens reçus pendant au moins cinq ans. Quant aux entreprises, elles bénéficient d'une exonération de 75 % à condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins quatre

qui permettrait de constituer une garantie de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d'une exonération de 80 % de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 20 millions d'euros. Ce dispositif existe notamment en Allemagne, en Italie et en Suisse. La parole est à M. Vincent

agricoles et viticoles familiales en allégeant la fiscalité de donations des successions. La parole

d'une réforme fiscale majeure, qui aura un impact de 18 milliards d'euros répartis sur la durée de la mandature, ce qui représente le quart de l'impôt sur le revenu. Nous sommes tous conscients que l'on n'engage qu'une grande réforme fiscale majeure par mandature. La voilà.

la taxe d'habitation par une ressource fiscale conforme à la réalité économique et assurée d'une dynamique. En ce qui concerne les communes, ce remplacement sera assuré par le basculement de la taxe foncière sur les propriétés

suite du débat. Pour les départements et les agglomérations, le choix retenu est celui de la TVA, qui assure une dynamique égale pour tous, alors que, si vous regardez la géographie de la France et ses effets économiques, vous comprenez qu'une grande partie des départements français seraient à terme perdants s'ils conservaient la ressource du foncier bâti qui ne sera pas dynamique dans les régions en affaiblissement,

lesquelles connaissent des variations démographiques beaucoup plus amples que celles des départements, il sera judicieux de prévoir à terme une prise en compte de la dynamique démographique des agglomérations dans le calcul de l'attribution de leur part de TVA. Le choix du calendrier

que ce que fixe le Gouvernement pour mener cette réforme d'ampleur, sans que cela ait d'incidence pour le contribuable, puisqu'il n'est pas question de remettre en cause la suppression de la taxe d'habitation. Le Gouvernement nous rétorquera que ce décalage n'est pas acceptable, pis, que c'est une mesure dilatoire ! Dans le même temps, il propose de ne réviser les valeurs locatives des locaux d'habitation qu'en ... Quand on sait l'importance de la distorsion de richesses imposée par la non-actualisation des valeurs locatives, on ne peut que déplorer ce calendrier. Pour voter cette réforme en toute connaissance de cause, avancer sur certains sujets centraux, qui nécessiteront du temps d'analyse et de concertation : je pense avant tout à la question de la péréquation. Ce travail est vital et ne doit pas être mené à la va-vite. Il est vital, parce que tout le reste de l'édifice financier local n'a plus de bases tangibles : la fiscalité est régulièrement réformée, souvent sans que les élus locaux le demandent les dotations sont dépassées, mais leur réforme n'est visiblement pas pour demain ... Restent les dotations et les fonds de péréquation qui, eux aussi, souffrent d'indicateurs souvent obsolètes. La suppression de la taxe d'habitation et la réforme du financement des collectivités territoriales qu'elle entraîne doivent être l'occasion de s'y pencher. Ce travail ne doit toutefois pas être mené au pas de charge, sous peine de se solder par un énième mécanisme de neutralisation des effets de la réforme, comme on en connaît tant. Nous nous y attellerons dès le début de l'année prochaine avec les rapporteurs spéciaux, pour tenter de trouver des critères et les indicateurs de péréquation plus justes, plus contemporains et plus adaptés à la diversité de nos territoires. Nous sommes à un carrefour, qui nécessite également de s'interroger sur la gouvernance globale des finances locales, en particulier sur leur encadrement par les contrats de Cahors. La libre administration des collectivités territoriales, clef de voûte de notre fonctionnement, est mise à mal par ces contrats. La réforme qui nous est proposée aujourd'hui par le Gouvernement doit donc être mise en perspective : un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales ne peut être mis en oeuvre sans que l'on revoie les règles actuelles d'encadrement et de gouvernance des finances locales.

une perte de recettes fiscales par une nouvelle recette fiscale et on garantit ainsi aux trois niveaux de collectivités une ressource pérenne et dynamique. Les communes retrouveront

sur les propriétés bâties et retrouver une part d'impôt national. Évidemment, il en résulte une perte d'autonomie fiscale pour les départements, mais vous savez ce que je pense de l'autonomie fiscale

plus ! Quel maire acceptera de construire du logement, d'accueillir de nouveaux habitants et de n'avoir aucune recette fiscale en retour ? C'est à cela que nous allons aboutir.

-qu'une allocation de compensation versée par l'État après la suppression ou l'exonération partielle d'une taxe relevait d'une ressource propre et participait à l'autonomie financière. La décision du 28 décembre 2019 peut faire l'objet de débats, mais elle pose aujourd'hui

les communes. Les masses sont importantes. Il s'agit de compenser aux communes 16 milliards d'euros de recettes de taxe d'habitation sur les résidences principales. Je rappelle que nous n'exonérons pas les résidences secondaires Nous avons fait le choix d'affecter aux communes la taxe foncière des propriétés bâties des départements, qui représente 15,1 milliards d'euros. L'écart de 900 millions d'euros sera

Nous avons fait ce choix, car la TVA, la taxe foncière sur les propriétés bâties et les frais de gestion sont des flux financiers qui transitent par le compte d'avance entre l'État et les collectivités. Cela nous garantit la nature fiscale des recettes de compensation.

à la hausse en termes de recettes ou de dépenses. Le fait que le FNGIR le soit pose aujourd'hui un certain nombre de difficultés, notamment pour des communes qui sont contributrices alors que leur situation économique et sociale s'est objectivement dégradée. Nous savons d'expérience que le potentiel fiscal des dégradée. Nous savons d'expérience que le potentiel fiscal des collectivités est un outil extrêmement fragile. Nous avons tous en tête l'année 2018. Elle a été la première année

le potentiel fiscal de 2018 a été calculé sur la base des derniers éléments connus, c'est-à-dire l'exercice 2017, qui était le premier exercice dans le cadre des nouveaux périmètres de l'intercommunalité. Dans la mesure où le potentiel fiscal d'une commune tient compte d'indicateurs socio-économiques de la commune, mais aussi de l'intercommunalité d'appartenance, des communes rurales appartenant à des intercommunalités rurales ayant rejoint des intercommunalités plus urbaines et, surtout, plus industrielles ont vu leur potentiel fiscal augmenter et ont automatiquement perdu le bénéfice de la DSR cible. En outre, en 2015, le CFL a inventé un mécanisme de sortie en sifflet de la DSU et de la DSU cible pour les communes les plus urbaines, mais n'a pas mis en place de mécanisme de sortie en sifflet pour la DSR cible. Cela s'est traduit par un quitte ou double en termes de DSR cible. Les communes qui sont sorties de la DSR cible y ont perdu brutalement, avec des baisses extrêmement fortes de dotations. Nous ne voulons pas connaître le même phénomène en 2022. La modification du panier de recettes fiscales des collectivités en 2021 se traduira mécaniquement par une modification de leur potentiel fiscal en 2022. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé devant votre délégation aux collectivités territoriales voilà quelques semaines, devant le Comité des finances locales, devant l'Assemblée nationale et, avant-hier, devant l'assemblée générale du Congrès des maires de France que l'on puisse mettre à profit les six premiers mois de l'année 2020

sur une nouvelle modalité de calcul du potentiel fiscal dans les six mois, nous aurions la possibilité d'introduire une mesure de neutralisation des effets de la modification du panier fiscal sur le potentiel fiscal, afin d'éviter que la modification

de locaux d'habitation. Quand on compare ces chiffres, on peut imaginer qu'il nous faille la durée que nous affichons entre 2020 et 2024 ou 2025, avec application en 2026. Je souhaite répondre à M. Dallier

blanche ». La rédaction actuelle de l'article aboutit à constater un décalage de TVA d'une année dans la prise en compte de l'évolution de TVA servant de référence et à perdre, en 2021, pour les collectivités concernées, une année d'évolution de la TVA substitutive de recettes. Nous proposons d'y remédier par cet amendement.

il va écouter, subir, être battu régulièrement, puis il fera rétablir tout ça à l'Assemblée nationale, tranquillement. Donc, restons sereins et calmes sur le devenir de tous ces amendements.

souvenez-vous de ce qu'il s'est passé lorsque le Gouvernement n'a pas écouté le Sénat sur la fiscalité de l'énergie. Souvenez-vous d'un certain nombre de sujets sur lesquels le Gouvernement, trop sûr de lui, a lourdement payé cette

Le scrutin est ouvert.

La taxe d'habitation est maintenue pour les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Elle est donc maintenue pour les organismes privés non lucratifs gérant des activités sanitaires, sociales et médico-sociales,

En 1999, un périmètre dit PIG a été défini afin de délimiter les terres polluées autour de l'usine. Les habitants des communes concernées subissent un préjudice important : ils ne peuvent plus construire comme ils le veulent cultiver leurs terres et enregistrent une moins-value de leur habitation. Du fait de ces préjudices, une disposition a été votée dans la loi de finances rectificative du 29 décembre 2016, permettant un abattement de 50 % de la taxe foncière pour tous les propriétaires touchés et prévoyant une compensation à l'euro près par l'État. Les élus des communes concernées et l'EPCI ont voté cet abattement pour qu'il puisse être applicable en 2018, mais la compensation de l'État n'est jamais arrivée du fait d'une impossibilité juridique. Cet amendement vise à rendre enfin possible cette compensation. Quel

trouve injustifié et particulièrement maladroit, pour une différence qui va peser une centaine de millions d'euros, d'expliquer dès le début de la discussion que l'on n'appliquera pas la revalorisation normale, sur laquelle le Parlement s'est prononcé de longue date, qui est raisonnable et qui correspond à la réalité économique.

comme le prévoit actuellement l'article, pour déterminer le montant de la perte de taxe d'habitation à compenser aux communes et aux EPCI à fiscalité propre.